Jamais dans l’histoire contemporaine un peuple n’a été aussi méthodiquement isolé, affamé, bombardé, privé d’accès aux soins et aux secours ! Gaza est aujourd’hui le théâtre d’une catastrophe humanitaire totale, sans précédent, qui a été rendue possible par l’inaction de la communauté internationale et le silence complice de nos grandes puissances C’est la première guerre moderne durant laquelle aucun couloir humanitaire n’a été mis en place, la première guerre moderne durant laquelle des blessés graves ne peuvent être évacués, la première guerre moderne durant laquelle des enfants meurent de faim à quelques mètres d’entrepôts pleins d’aide humanitaire volontairement bloquée, guerre moderne durant laquelle des médecins de retour du théâtre des opérations entament des grèves de la faim pour exiger un cessez le feu et un corridor humanitaire. Cette réalité interroge notre conscience collective. Quand des femmes accouchent au sol, sans anesthésie, quand des chirurgiens opèrent à la lumière des téléphones portables, sans eau, sans médicaments, quand l’odeur de la mort remplace celle de la vie, ce

! Chaque jour qui passe sans cessez le feu, sans aide, sans voix pour crier son désarroi face à la réalité est une trahison de nos valeurs fondamentales et de la dignité humaine ! Dans ce contexte, il est temps de passer des discours aux actes. si, comme l’affirme le Président de la République, notre pays est opposé à toute annexion de Gaza et de la Cisjordanie, la France doit soutenir le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et reconnaître sans tarder l’État de Palestine, unique levier pour imposer enfin le respect du droit international et stopper le génocide. Monsieur le ministre, notre pays compte t il prendre ses responsabilités ? Entend il exiger un cessez le feu immédiat, l’ouverture d’un corridor humanitaire, le respect des décisions des instances internationales ? Enfin, quand reconnaîtrez vous l’État de Palestine ?

a parlé ! … pour apporter huit tonnes de fret humanitaire, se rendre au chevet des blessés palestiniens, qui sont aujourd’hui soignés en Égypte, et aller à la rencontre des acteurs humanitaires qui continuent courageusement de tenter d’apaiser les souffrances du peuple palestinien.

stabilité à l’ensemble de la région. C’est dans cet esprit que nous agissons. C’est dans cet esprit que le Président de la République s’est rendu en Égypte ces deux derniers jours. Monsieur le ministre, quand le droit s’efface devant la force, quand la dignité humaine devient une variable d’ajustement diplomatique, c’est tout l’ordre international qui vacille ! Soyez fidèles à ce que la France a longtemps été et à ce qu’elle devrait rester ! La

Républicains. Monsieur le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, « les mots “droits de douane” sont les plus beaux mots du dictionnaire ». C’est ce que déclarait Donald Trump dans ses meetings lorsqu’il était candidat à la présidence des États Unis.

comment ne pas s’interroger sur l’impréparation de l’Europe ? Après tout, Donald Trump ne fait que ce qu’il avait annoncé ; comment ne pas le reconnaître ? Nous, Européens,

il n’y a qu’à consulter les résultats des sondages d’opinion réalisés aujourd’hui aux États Unis pour s’apercevoir que les Américains sont parfaitement conscients de l’impact que ces décisions désastreuses vont avoir sur leur pouvoir d’achat. Face à cette situation, nous disons bien évidemment que ces décisions sont mauvaises et nous espérons vivement qu’elles puissent être revues. Nous disons également que nous ne les avons pas provoquées et que, si le président Trump ne revenait pas dessus, nous nous tenons prêts, qu’Européens, à riposter en mobilisant toute la palette des instruments à notre disposition, qu’ils soient tarifaires ou non tarifaires. C’est du reste tout l’enjeu de la première salve de contre mesures qui ont été adoptées au

l’application d’une deuxième salve de mesures. En attendant, le Président de la République, avec le Premier ministre et plusieurs membres du Gouvernement, a réuni les filières concernées dès jeudi dernier. Hier, c’est le ministre de l’industrie qui a convoqué le Conseil national de l’industrie ; aujourd’hui, c’est le ministre de l’économie et des finances

d’information pour revoir les nouveaux paradigmes du commerce international. du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, Là où Donald Trump passe, le commerce trépasse ! Depuis six heures ce matin, des droits de douane additionnels s’appliquent au monde entier ou presque. Pour la France, pour l’Union européenne, le tarif est de Cette guerre commerciale apporte une mauvaise réponse à un mauvais diagnostic. Il s’agit d’un mauvais diagnostic, parce que le président Trump veut résorber de prétendus déficits commerciaux, alors qu’il ne prend en compte que les biens et pas les services, secteur dans lequel les États Unis sont largement excédentaires. mauvaise réponse, parce que nos économies sont désormais totalement interdépendantes. À titre d’exemple, les entreprises françaises emploient 700 000 salariés aux États Unis quand les entreprises américaines emploient 400 000 salariés en France.

des produits de luxe, des cosmétiques, des produits pharmaceutiques… Heureusement, l’Union européenne n’est plus l’idiot du village global, ouvert à tous les vents ; elle s’est armée et réarmée en matière commerciale. Monsieur le ministre, plusieurs questions se posent.

La parole est à M. Pierre Jean Rochette, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. Monsieur le président, permettez moi d’associer mes trois collègues sénateurs de la Loire à ma question. Monsieur le ministre

très importante, celui de la production d’armes dans la région stéphanoise. En revanche, je tiens à le préciser ici, aujourd’hui, l’entreprise n’a pas de contrat stratégique en lien avec nos enjeux nationaux de défense.

Ils renchérissent aussi le coût de la vie sur l’archipel, qui est totalement dépendant de l’acheminement maritime depuis l’Hexagone ou le Canada. Ensuite, elle est structurelle : nos infrastructures de transport sont à bout de souffle. Les quais des ports d’État, à Saint Pierre comme à Miquelon, menacent de s’effondrer. Et nous avons récemment appris, à l’Assemblée nationale, qu’aucun financement n’est prévu avant 2027…

En 2019, le Gouvernement avait promis un fonds d’innovation et de diversification pour en compenser les effets. Nous l’attendons toujours… Monsieur le ministre, ma question est simple

; et, hier, ce sont des voix qui s’élèvent pour faire de l’archipel un centre de rétention administrative… Il convient de rappeler que tous les territoires ultramarins sont membres à part entière

je relève que, après les déclarations fracassantes dans le Bureau ovale, Saint Pierre et Miquelon a été retiré du décret présidentiel introduisant les droits de douane que vous Ensuite, je vous assure que tous les territoires de la République seront pris en compte dans les préconisations qui seront faites par la France à la Commission européenne, pour que celle ci ajuste sa réponse et, éventuellement, sa réplique, avec, à l’esprit, d’obtenir le retrait de ces droits de douane et, en tout état de cause, celle de défendre les filières, comme l’évoquait à l’instant le ministre de l’économie et des finances. Par ailleurs, et sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, ici, au Sénat, vous avez évoqué le Ceta

La parole est à M. Christian Redon Sarrazy, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. de l’Europe et des affaires étrangères, les conséquences potentiellement dévastatrices des taxes annoncées par Donald Trump inquiètent à juste titre le monde économique et nos compatriotes. Selon les économistes, la stratégie de négociation « zéro pour zéro » de la Commission européenne sera préjudiciable aux intérêts de la France et de nos filières les plus exposées : l’aéronautique, l’automobile, les vins et spiritueux notamment. Une telle réponse profitera avant tout à l’Allemagne et à l’Italie compte tenu de leurs excédents commerciaux. Alors, quelles options nous reste t il ? Le président américain ne reviendra pas sur sa décision.

La bonne réponse consiste en une relocalisation de certaines filières et en la mise en place de droits de douane ciblés, accompagnés de ce que nous demandons depuis longtemps, une stratégie de planification industrielle qui renforcera notre souveraineté et améliorera notre balance commerciale. Elle protégera aussi le marché européen et français de l’ajustement stratégique que la Chine, après la fermeture du marché américain, ne va pas manquer d’opérer pour déverser ses surcapacités sur le vieux continent. Allez vous défendre cette stratégie auprès de la Commission européenne, seule entité capable de protéger les Français et de permettre à la France et à l’Europe de reprendre en main leur destin économique ? Pour une fois, soyons des pionniers en envisageant une nouvelle adaptation, et ne partons

de rappeler que nous ne devons pas nous contenter de répondre à l’administration américaine. Nous devons nous poser des questions sur nous mêmes. Nous nous apercevrons que le marché unique n’a sans doute jamais été aussi important pour permettre à nos entreprises de se diversifier. Les barrières qui se dressent entre les pays de l’Union européenne représenteraient des droits de douane d’environ 45 %.

comme vous l’avez dit, nous entrons dans une période de guerre commerciale, nous devons nous y préparer en gagnant en compétitivité et en retirant la chape de plomb qui empêche les entreprises françaises

pour être en mesure non pas seulement de défendre nos intérêts, mais aussi, dans cette période de tension commerciale, de gagner des parts de marché. Monsieur le ministre, que cela soit dit, les Français n’ont pas à assumer les conséquences budgétaires du diktat américain, alors même que nos grands groupes veulent continuer, au mépris de tout patriotisme économique, d’investir aux États Unis pour contourner les droits de douane ils refusent explicitement de soutenir notre économie et font preuve d’une indifférence totale aux inquiétudes des Français face à la crise qui s’annonce. Nous attendons du Gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour éviter l’effondrement de certaines filières et faire en sorte que le pouvoir d’achat des Français ne soit pas une nouvelle fois amputé par des hausses de prix.

Vous avez énoncé clairement et avec force que l’accord de Nouméa constituait le socle intangible sur lequel la négociation devrait se fonder. Vous avez également confirmé à maintes reprises que le droit à l’autodétermination du peuple colonisé,

Tu saurais où se trouve la porte si tu avais aidé à construire la case ! » La trajectoire politique d’émancipation et d’évolution institutionnelle engagée depuis 1983

Dès le 29 janvier, j’ai écrit à toutes les formations politiques – vous avez lu le texte, vous en avez cité des passages – pour leur proposer d’ouvrir des discussions afin de trouver un accord politique

Dès le mois de février, des réunions se sont tenues, à Paris, puis à Nouméa, où le ministre d’État s’est rendu à deux reprises. Un premier document d’orientation a été mis sur la table, puis un projet d’accord, dont toutes les parties

selon une méthode que j’ai voulue respectueuse de chacun et qui s’intègre dans une histoire marquée par les accords de Matignon Oudinot, puis de Nouméa. La question de l’autodétermination est évidemment centrale. Elle a été rappelée par tous les aspects du droit : elle est reconnue par les textes internationaux, dont la Charte des Nations unies, mais aussi par notre Constitution, en son article 53.

Les options sont sur la table, vous les connaissez, et je sais votre aspiration à une souveraineté pleine et entière de la Nouvelle Calédonie. Le ministre d’État a déjà annoncé qu’il reviendrait à Nouméa à la fin du mois d’avril pour poursuivre ces discussions.

En zone rurale, ce chiffre s’élève à deux sur trois, contre seulement un sur quatre en zone urbaine : voilà un révélateur brutal de la fracture territoriale qui s’installe progressivement. Pourtant, l’engagement des élus ne faiblit pas. Souvent au prix de leur vie personnelle ou professionnelle, ceux ci ont fait le choix altruiste de servir les autres, de servir la République.

à eux. Ils demandent une reconnaissance plus juste de leur engagement par le biais d’une indemnisation digne et d’une adaptation cohérente du calcul de leur retraite pour qu’il tienne compte de leur choix de faire primer leur engagement citoyen sur leur carrière professionnelle.

Madame la ministre, en cette période clé de constitution des listes électorales, à quelle date cette proposition de loi sera t elle inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ? Quelles mesures concrètes le Gouvernement entend il y intégrer pour envoyer un message fort et clair à nos élus locaux ? La parole

Depuis, les provocations se multiplient : blocages, occupations, prières en plein campus, invectives publiques contre une direction accusée de racisme et d’islamophobie… Le 1 avril, un nouveau cap a été franchi : quinze militants cagoulés ont violemment interrompu le cours du professeur Fabrice Balanche en l’injuriant, le menaçant et le traitant de sioniste et de génocidaire. Certes, vous avez affiché votre soutien. Pourtant, la salle est toujours occupée. Les intimidations continuent. L’idéologie qui y est professée est antifrançaise, radicale et violente ! Madame la ministre d’État, nous voyons nos universités devenir des zones de non droit. Est ce tolérable ? Est ce acceptable ?

de façon respectueuse. C’est dans cette logique que je défendrai toujours les libertés académiques et la liberté d’expression. Vous le savez, l’université a immédiatement réagi en accordant la protection fonctionnelle

de nouveau cette agression ; fort bien ! Samedi, Jean Michel Blanquer vous a lancé un appel à agir. Interrompre un cours est une attaque frontale contre les libertés académiques, et celui du professeur Balanche n’a pas été interrompu par hasard. Il a été ciblé : ciblé pour ses travaux sur le Moyen Orient ; ciblé parce qu’il refuse de céder à l’intimidation intellectuelle. Des idéologues gauchistes et islamistes l’ont pris pour cible, comme ils l’ont fait hier avec Gilles Kepel, Bernard Rougier ou Florence Bergeaud Blackler. Jusqu’à quand laisserons nous faire ? Madame la ministre, il faut agir maintenant, fermement, clairement, courageusement ! Vous devez exiger l’évacuation des locaux et l’exclusion des agresseurs. Vous devez vous porter partie civile, comme vous venez de Le ministère de l’intérieur protège ses policiers ; il est temps que le ministère de l’enseignement supérieur protège ses professeurs ! Car sans liberté académique, il n’y a plus d’université !

des procès ont eu lieu, des travailleurs sociaux ont alerté, des enfants ont témoigné. D’autres ne le peuvent plus. Personne ne peut ignorer l’état de la protection de l’enfance et le sort des 400 000 enfants accompagnés, parfois, protégés, mais pas toujours. L’écart entre ce qui est dit et su et la réalité de l’action est immense.

Quand obtiendrons nous enfin une loi pluriannuelle des moyens alloués à la protection de l’enfance pour tracer de vraies perspectives ? Qu’avez vous fait du rapport sur le travail social ? Ne pas renforcer les métiers du lien, c’est creuser le gouffre de la protection de l’enfance. Aujourd’hui, il faut agir Chacun de ces 400 000 enfants est une figure républicaine à l’égard de laquelle notre responsabilité est immense. Ces enfants tiennent, parfois sous les coups, souvent sous les dominations ou le déni. Certains ne tiennent pas.

Dans la nuit du 3 au 4 avril dernier, 830 kilos de cocaïne ont encore été interceptés. En Guyane, le dispositif d’interception des mules a fait diminuer radicalement les passages. Toutefois, il faut voir dans ces prises le corollaire de l’augmentation de la production. Les chiffres sont alarmants et suscitent de vives inquiétudes pour les territoires français de la Caraïbe, qui sont particulièrement exposés en raison de leur position géographique. Il y a deux semaines, une chaîne de télévision diffusait un reportage montrant, en Guadeloupe,

Localement, l’inquiétude que nous partageons est de voir la ville tomber aux mains des trafiquants, ce qui offrirait un point de passage facilité à la drogue et aux armes. nous ne pouvons pas rester inactifs. La part des mineurs dans les rangs des gangs est évaluée à 30 %. Bien sûr, nous ne pouvons pas demander à l’armée d’intervenir contre des enfants.

remercie, monsieur le ministre. Aider Haïti, c’est aussi aider les outre mer caribéens et je sais que je peux compter sur votre détermination et sur celle de la France.

Je sais que le ministre de l’économie s’apprête à recevoir les représentants de ces secteurs exportateurs dans quelques minutes. Ensuite se pose la question de l’impact pour nos finances publiques. Comment comptez vous faire face au choc supplémentaire que ces droits de douane induiront pour nos finances publiques,

permanent. Il est devenu un phénomène social majeur, qui contribue en grande partie à la dégradation des apprentissages et, plus largement, de la réussite scolaire. À la rentrée de septembre 2024, une expérimentation de l’interdiction effective du téléphone portable au collège a été lancée.

elle est expérimentée dans une centaine de collèges depuis la rentrée de 2024, et tous les retours sont très positifs. On observe notamment une amélioration du climat scolaire et le

En 2024, 2 800 enfants ont perdu la vie avant leur premier anniversaire. Cette dégradation catastrophique frappe particulièrement les départements les plus pauvres et les départements ruraux,

pour assurer une bonne répartition territoriale. En cinquante ans, 75 % de nos maternités ont disparu : nous sommes passés de 1 369 maternités publiques en 1975 à 457 en 2024. en 2024. Or ces fermetures – chacun le sait – augmentent le risque de morbidité et de complications pour la mère comme pour l’enfant. Madame la ministre, pouvons nous continuer à sacrifier l’accès aux soins des femmes et des enfants sous prétexte de rationalisation ? Devons nous poursuivre la fermeture des maternités réalisant moins de 1 000 naissances par an et laisser tant de femmes accoucher sur les routes ?

que je prends devant vous, à la demande de M. le Premier ministre. m’interroge : devons nous continuer, dans nos territoires, à être maltraités à la naissance, ignorés une fois devenus adultes, puis abandonnés lorsque nous devenons seniors et approchons de la fin de notre vie ? Doit on continuer à fermer les yeux sur la tiers mondisation de notre système de santé ? La parole est à M. Christophe André Frassa, pour le groupe Les Républicains. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cela fait aujourd’hui près de quatre ans que notre compatriote Paul Maillot, condamné à vingt ans de travaux forcés, purge sa peine dans des conditions innommables à Madagascar.

tant le caractère arbitraire de la détention de M. Maillot est devenu une évidence. Les Nations unies l’ont confirmé dans un récent avis en demandant sa libération immédiate. Paul Maillot représente aujourd’hui un moyen de pression dans les relations bilatérales entre la France et Madagascar. Il ne doit pas en être l’otage. Sa double nationalité, souvent invoquée par les Malgaches pour justifier l’absence de réponse favorable à son sujet, n’est qu’un argument de façade – convenons

doit apporter son concours à l’application de l’avis de l’ONU en demandant la libération de Paul Maillot. Sa fille aînée, que j’ai eu l’occasion de rencontrer à de nombreuses reprises et qui se trouve cet après midi en tribune, est éreintée par cette situation, en particulier par la responsabilité de la survie de son père, depuis la France. Les Malgaches souhaitent rééquilibrer nos relations bilatérales : soit. Cela doit passer par le retour en France de Paul Maillot dans les plus brefs délais.

la situation de Paul Maillot est suivie de très près par les services de mon ministère et par le Gouvernement tout entier, sous l’autorité du Premier ministre.

Par ailleurs, nous entretenons un dialogue soutenu avec les autorités malgaches, dans le cadre de la coopération judiciaire qui lie nos deux pays. Les conditions de détention de Paul Maillot sont pour nous source de vives inquiétudes, et nous plaidons pour leur amélioration. Enfin, nous restons aux côtés de la famille de Paul Maillot. Sa fille a été reçue par mon cabinet le 24 février dernier et nous veillerons à maintenir le dialogue avec les différents membres de sa famille.

en tentant d’obtenir l’amélioration de leurs conditions de détention et leur libération. Nous sommes également aux côtés de leur famille, en leur apportant tout le soutien moral que nous pouvons leur donner. Monsieur le ministre, il est temps de faire un peu plus que du soutien moral… Oui ! Les autorités malgaches utilisent Paul Maillot comme un otage dans leurs relations bilatérales

en 2022, le Président de la République annonçait, au titre du renforcement de la sécurité intérieure et de la présence de l’État, la création de 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Il s’agissait de répondre à de fortes attentes en luttant contre les déserts sécuritaires, en faisant revenir durablement la force publique dans les territoires, notamment les territoires ruraux.

Pourtant, plusieurs signaux d’alerte remontent du terrain. Dans de nombreuses communes, les élus ont fait leur part du chemin : délibérations votées, crédits mobilisés, bâtiments rénovés ou du moins identifiés. Mais les effectifs attendus ne sont pas là.

tous attendent que la promesse présidentielle soit tenue. Pouvez vous nous indiquer où en est concrètement la programmation, quand les effectifs seront déployés et si tous les engagements seront honorés dans les délais annoncés ? La parole est à M.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai l’honneur de vous demander de reconnaître la responsabilité de l’État dans les préjudices moraux et sanitaires subis par les populations de Guadeloupe et de Martinique, qui ont été exposées, pendant deux décennies, à un produit phytosanitaire toxique : le chlordécone. Il est des scandales si profondément enracinés qu’ils traversent les décennies sans perdre leur capacité En effet, de 1972 à 1992, l’État a autorisé la mise sur le marché de ce produit destiné à lutter contre le charançon de la banane, oubliant l’avertissement donné, dès 1968, par la Commission interministérielle d’étude de l’emploi

Cette pathologie n’est malheureusement pas la seule à affecter la population. Ainsi, une exposition chronique à la pollution rémanente par le chlordécone est susceptible non seulement de réduire la durée de la grossesse, mais également de provoquer un accouchement prématuré, ce qui peut entraîner de graves complications chez l’enfant, voire son décès. L’exposition L’exposition des parents à cette pollution rémanente est associée chez l’enfant à des troubles neurodéveloppementaux, au développement de leucémies et de tumeurs cérébrales, mais aussi à l’apparition d’une fente labio palatine, appelée communément bec de lièvre, ou d’un hypospadias, une malformation sexuelle. Ces maladies et ces troubles du développement sont attestés et validés par la science. Le cancer de la prostate lié à une surexposition au chlordécone a été inscrit, le 22 décembre 2021, au tableau des maladies professionnelles. Une étude de cohorte, l’enquête Ti Moun, menée depuis 2004, a permis d’observer que l’exposition chronique au chlordécone de la femme enceinte est associée de manière significative à une réduction de la durée de la grossesse. Ainsi, le risque de prématurité est accru pour les femmes présentant des concentrations de chlordécone dans le sang supérieures à 0,52 microgramme par litre. En outre, des travaux sur le neurodéveloppement de l’enfant, publiés en 2022, démontrent qu’une exposition pré et postnatale au chlordécone pourrait affecter le développement cognitif et le comportement de l’enfant. Dans un arrêt récent, le 11 mars le 11 mars 2025, les juges de la cour administrative d’appel de Paris ont reconnu qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques, des pathologies graves sont susceptibles de se développer à la suite d’une exposition chronique au chlordécone : cancer de la prostate et sa récidive chez l’homme ; prééclampsie chez la femme enceinte ; troubles du développement chez l’enfant à naître et cancers pédiatriques. la cour administrative d’appel a condamné l’État à indemniser une dizaine de requérants, qui demandaient réparation du préjudice d’anxiété subi du fait de leur contamination au chlordécone. Ma proposition de loi vise donc à permettre à l’ensemble de la population de Guadeloupe et de Martinique d’obtenir réparation du préjudice d’anxiété subi du fait de son exposition au chlordécone sans avoir à introduire de recours devant le juge administratif.

sont remplies et d’accorder les indemnisations sollicitées. C’est donc à regret que j’ai appris que la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable n’avait pas adopté ce texte, estimant qu’il n’était pas suffisamment équilibré. Cet argument est difficile à entendre pour les personnes exposées au chlordécone depuis des dizaines d’années et qui le seront encore longtemps. Cela paraît d’autant plus injuste que le présent texte fixe précisément, selon le consensus scientifique international, les conditions de la réparation. L’article 1 vise ainsi à reconnaître la responsabilité de l’État pour les préjudices causés par l’utilisation du chlordécone et subis par les populations antillaises et à fixer le principe d’une indemnisation de ces populations ainsi que l’obligation d’organiser une campagne de prévention à l’échelle nationale. J’insiste sur la responsabilité de l’État dans son arrêt du 11 mars dernier, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que « l’État a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard des requérants qui invoquent leur exposition à la pollution rémanente par le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe ».

L’article 2 tend à fixer les conditions dans lesquelles les populations peuvent obtenir l’indemnisation prévue à l’article 1 en imposant au demandeur la charge de la preuve de la preuve pour le lieu et la durée de séjour, ainsi que les préjudices indemnisés au titre de la présente proposition de loi. Par ailleurs, le même article 2 prévoit que la liste des pathologies résultant d’une exposition au chlordécone, reconnues comme telles par la communauté scientifique internationale, soit fixée par décret. Il a également pour objet de limiter le délai de recours à l’indemnisation à six ans à compter de la promulgation du présent texte ou du développement d’une pathologie liée à l’exposition au chlordécone.

De tels critères correspondent au consensus scientifique international en la matière, rappelé par la cour administrative d’appel de Paris, contrairement à ce qu’a indiqué la commission lors de ses travaux. L’article 3 tend à ce que l’indemnisation soit versée sous forme de capital et déduite d’éventuelles réparations déjà perçues par le demandeur. Cette disposition permet de répondre à la critique présentée par la commission, qui s’inquiétait du fait qu’un travailleur ayant déjà bénéficié d’une réparation au titre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) puisse de nouveau y prétendre au titre de la présente proposition de loi. l’article 4, je propose la création d’une autorité administrative indépendante, le Comité d’indemnisation des victimes du chlordécone (Civic), chargée d’examiner les demandes d’indemnisation présentées par les populations de Guadeloupe et de Martinique. Cet article a aussi pour la victime demandant une indemnisation si les critères fixés par le législateur sont réunis. Sur ce point, je souhaite insister sur la nécessité pour le Civic de demeurer une autorité administrative indépendante, afin de se prémunir de tout risque d’impartialité.

que les indemnités versées par le Civic soient affranchies de l’impôt. Enfin, l’article 6 donne au Civic les moyens de mener à bien sa mission de service public

refuser ce texte, ce serait prolonger la rémanence non plus du pesticide, mais de l’indifférence. Je souhaite que nous prenions nos responsabilités, ici et maintenant, pour réparer, pour reconnaître, pour reconstruire.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans ses, le général de Gaulle exprimait, avec gravité et hauteur de vue, la mission fondamentale de l’État en ces termes, désormais inscrits dans notre mémoire collective : « aussi l’État, qui répond de la France, est il en charge, à la fois, de son héritage d’hier, de ses intérêts d’aujourd’hui et de ses espoirs de demain

Ce texte vise à répondre, avec responsabilité et dignité, à une situation douloureuse : celle des dommages subis par les populations des Antilles françaises à la suite de l’utilisation prolongée du chlordécone. Je tiens à saluer très sincèrement l’engagement de son auteur, notre collègue Dominique Théophile. Voilà plusieurs années que le chlordécone est un sujet particulièrement cher au Parlement. Ainsi, depuis le début des années 2000, pas moins de cinq initiatives parlementaires, essentiellement issues de l’Assemblée nationale, et cinq rapports d’information ont enrichi le débat public sur ce sujet si sensible.

des milieux aquatiques et de la faune et de la flore de Guadeloupe et de Martinique. Sur un sujet voisin, qui n’est pas sans présenter des similitudes avec les enjeux soulevés par le texte que nous examinons, notre collègue Nicole Bonnefoy avait souligné, à la faveur de la mission commune d’information sur les pesticides, présidée par Sophie Primas, les difficultés environnementales et sanitaires que posait l’utilisation de nombreux pesticides. Je salue la qualité de sa réflexion, ainsi que son engagement. Sans aborder exclusivement le cas du chlordécone, notre collègue Bonnefoy mettait ainsi en avant, sans le nommer, un besoin de reconnaissance et d’indemnisation des victimes exposées à ces substances profondément néfastes à la santé humaine.

la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, apporte une réparation forfaitaire aux personnes exposées professionnellement aux pesticides et bénéficiant d’une reconnaissance de maladie professionnelle reconnue par l’assurance maladie. Il indemnise également les parents de victimes exposées à des produits phytosanitaires ayant favorisé le développement de pathologies chez l’enfant. Si j’évoquais précédemment la proximité de ce fonds avec notre sujet du jour, c’était non seulement pour dresser un parallèle indemnitaire et thématique, mais également pour souligner que ce fonds est un premier point d’entrée sur le long chemin de l’indemnisation des victimes du chlordécone. Ces dernières peuvent en effet le saisir, afin d’obtenir réparation du cancer de la prostate, reconnu depuis 2021 comme maladie d’origine professionnelle en raison d’une exposition aux pesticides. Cette avancée, heureuse et récente, était d’autant plus nécessaire que cette pathologie est aujourd’hui la seule dont le lien causal avec l’exposition au chlordécone est scientifiquement établi, comblant ainsi un vide indemnitaire.

sans en contester l’économie générale, ni même le bien fondé. En effet, nous ne pouvons rester sourds aux demandes légitimes d’une population victime de cette contamination à grande échelle. Encore une fois, je veux saluer l’engagement remarquable de notre collègue Théophile. Mes travaux préparatoires de rapporteure m’ont conduite à entendre quatorze personnes, pour un total de huit heures d’auditions, dans des temps particulièrement contraints. Partie d’une feuille blanche, mon cheminement est le résultat de l’avis d’experts, d’acteurs institutionnels et de témoignages de victimes.

Tout naturellement, la commission joue son rôle en déposant un amendement tendant à préciser la portée de la responsabilité de l’État et à la circonscrire aux dommages sanitaires. Cette précision sémantique pourrait paraître anecdotique, mais elle revêt, en droit de la responsabilité et de la réparation,

le caractère certain, déterminé et direct du dommage. Nous avons également souhaité conférer au nouveau fonds un statut plus approprié que celui d’autorité administrative indépendante. Ce formalisme juridique se justifie en effet dans des situations de doute et de soupçon quant à la partialité supposée de l’autorité chargée de prendre des décisions. En l’espèce, mes auditions n’ont pas fait apparaître une telle défiance. C’est pourquoi j’ai déposé un amendement à l’article 4.

Les personnes que j’ai entendues, notamment les chercheurs et scientifiques, ont toutes insisté sur la nécessité d’approfondir la recherche sur les liens entre exposition au chlordécone et développement de pathologies. Alors que la relation entre expertise, science et prise de décision est plus que jamais prégnante, nos espérances se tournent vers la recherche. Seule la science peut valablement ouvrir un chemin crédible de réparation. L’article 2 du présent texte pose le principe d’une indemnisation large des victimes, sur la base d’une liste de pathologies établie après décret en Conseil d’État. Cependant, si personne ne conteste le principe d’une telle indemnisation, mes travaux ont fait apparaître un besoin de temps long, afin de ne pas comprimer l’irréductible temps de la science. Or, en l’état des connaissances scientifiques, je crains que le régime de réparation proposé dans le texte ne se limite à l’indemnisation du cancer de la prostate. J’achèverai mon propos en insistant sur l’importance de bâtir un régime d’indemnisation crédible et proportionné. Ce jalon est essentiel au rétablissement du lien de confiance qui unit la métropole à ses territoires ultramarins des Antilles. La parole

qui emporte des enjeux historiques, juridiques, sanitaires, sociaux et environnementaux, dont nous débattons cette après midi. Ce sujet n’est pas nouveau. Il est le fruit d’une époque et de pratiques tardivement, mais heureusement, révolues.

L’État doit y répondre en responsabilité, c’est à dire sans détour, en regardant le sujet en face, en le prenant dans sa globalité, tout en envisageant ses multiples facettes. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je voudrais commencer par saluer l’engagement du sénateur Dominique Théophile, comme celui de tous les parlementaires ultramarins, qui portent l’enjeu du chlordécone avec conviction depuis des années. Votre proposition de loi marque une nouvelle étape sur le chemin de la réparation des dommages liés à l’autorisation de cet insecticide toxique. Cette nouvelle étape porte d’abord sur la reconnaissance de la responsabilité de l’État.

Elle n’est plus à démontrer et a déjà été reconnue par des décisions de justice, ainsi que par le chef de l’État lui même dans son discours de septembre 2018, à Morne Rouge, en Martinique.

Dans ce cadre, la formulation proposée par Mme la rapporteure Nadège Havet, dont je salue l’important travail sur ce texte, me semble être tout à fait juste, à la hauteur des enjeux et de nature à rassembler. En effet, cette rédaction permet de bien reconnaître une responsabilité des pouvoirs publics, à une époque d’aveuglement collectif ayant conduit à continuer d’autoriser et d’utiliser le chlordécone, alors que d’autres territoires avaient cessé bien plus tôt

Depuis 2020, le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides a permis de dédommager les professionnels directement touchés. L’article 2 du texte permettra de renforcer les possibilités d’indemnisation de toutes celles et de tous ceux qui subissent un dommage sanitaire. C’est, encore une fois, juste et légitime.

Je salue l’important travail réalisé sur ce point par la rapporteure. La rédaction qu’elle propose permettra de mettre en œuvre concrètement ce nouveau dispositif, au bénéfice des victimes.

Notre méthode repose sur la prise en compte des travaux scientifiques, sur la concertation, sur l’écoute, sur le dialogue et sur la collaboration avec tous les acteurs locaux, partenaires essentiels, l’accompagnement des personnes concernées par cette pollution, car nous avons besoin de tout le monde pour sortir du risque chlordécone. Cela se traduit par des mesures très concrètes. Premièrement, pour tous les habitants,

ans, plus de 48 millions d’euros de fonds publics ont déjà été engagés, soit 22 millions de plus que les crédits consacrés au plan précédent, En tant que ministre de la santé, je compte m’appuyer sur cette mobilisation renforcée des moyens de l’État pour avancer sur deux points prioritaires. Le premier concerne la recherche pour l’amélioration continue des connaissances scientifiques, notamment sur la santé des femmes, et la dépollution des sols. À terme, ce volet devrait mobiliser 40 % des crédits de la stratégie. porte sur le dépistage et la prévention. La présence de chlordécone dans le sang n’est pas systématiquement dangereuse et, surtout, elle est réversible par des actions portant, notamment, il pour cela connaître son taux de chlordécone et savoir quelle action mettre en place. Depuis que je suis ministre, j’accorde toujours une attention particulière à la situation sanitaire de nos outre mer ; je serai attentif à ce que le dépistage du chlordécone devienne un réflexe en Guadeloupe et en Martinique afin d’accompagner plus vite et de manière toujours plus ciblée et personnalisée tous ceux qui en ont besoin. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, je respecte votre engagement et vous pouvez compter sur le mien pour réussir cette nouvelle étape dans l’histoire de la réparation des dommages liés au chlordécone. Il s’agit autant d’un sujet de santé publique et environnementale que d’une marque de considération pour les habitants de Martinique et de Guadeloupe. Je vous remercie et je reste à votre écoute.

car il s’agit aujourd’hui de réparer une injustice faite à des millions de nos compatriotes depuis des décennies. Comment ne pas entendre le cri de douleur de nos concitoyens de Martinique et de Guadeloupe, à 90 % intoxiqués dans leur chair et dans leur sang par ce pesticide rémanent, hautement toxique et cancérogène, qui empoisonne encore pour des centaines d’années les sols et les eaux des Antilles Comment ne pas entendre cette demande légitime de réparation d’un préjudice volontairement causé, dans l’un des derniers scandales d’État du XX siècle ? République : « La pollution à la chlordécone est un scandale environnemental, dont souffrent la Martinique et la Guadeloupe depuis quarante ans. […] Au fond, pendant des années, pour ne pas dire des décennies, nous avons collectivement choisi de continuer à utiliser la chlordécone, là où d’autres territoires avaient cessé beaucoup plus tôt. » s’agit donc bien d’un scandale d’État emportant des conséquences sanitaires, économiques, sociales et politiques qui ravagent encore le quotidien de nos compatriotes antillais. Pour rappel, le chlordécone est un pesticide organochloré utilisé dans les Antilles pour lutter contre le charançon du bananier et qui fut autorisé par l’État à partir des années 1970, et ce jusqu’en 1993. Pendant des décennies, les sols des Antilles ont été sciemment empoisonnés. Oui, sciemment, car la toxicité du chlordécone était connue des pouvoirs publics depuis 1968, soit quatre longues années avant l’autorisation officielle accordée par l’État en 1972. Cette autorisation, délivrée à titre dérogatoire, a été reconduite plusieurs fois par les autorités administratives et sanitaires pendant plus de vingt ce malgré la grande grève agricole de 1974 en Martinique, pendant laquelle les ouvriers ont exprimé leurs inquiétudes concernant le chlordécone, malgré l’incident survenu dans une usine en Virginie et l’interdiction du chlordécone dès 1976 aux États Unis, malgré les alertes répétées des scientifiques concernant le chlordécone, reconnu en 1979 comme perturbateur endocrinien probablement cancérogène. Au scandale d’État s’ajoute désormais un scandale sanitaire, car il s’avère que la Martinique détient le triste record mondial du taux d’incidence du cancer de la prostate. Par ailleurs, cet écocide affecte également l’activité économique et sociale dans le secteur agricole et de la pêche. Dès lors, en l’absence de réponse politique,

mais elle permet aussi des avancées en matière de reconnaissance des maladies professionnelles liées à l’exposition au chlordécone. En effet, en raison de la complexité des procédures d’indemnisation, seuls 150 dossiers ont été reçus à ce jour, pour 12 700 travailleurs en bananeraie. Aussi, dans la lignée des recommandations du dernier rapport sénatorial sur le chlordécone, notre groupe appelle également le Gouvernement à aller plus loin, en instaurant le dépistage systématique du cancer de la prostate dès 45 ans aux Antilles plus de moyens pour la recherche sur la dépollution des sols et sur le « zéro chlordécone » dans l’alimentation ; en communiquant plus avec les populations des Antilles et la diaspora de l’Hexagone sur la gratuité des tests sanguins en améliorant la formation des professionnels de santé par la création d’un institut spécifique dédié aux soins oncologiques, notamment pour les ouvrières agricoles, dont les cancers du sein ou de l’utérus ne sont toujours pas reconnus comme maladies professionnelles. En somme, mes chers collègues, en prenant un peu de recul, les choses sont simples : à l’instar d’autres scandales tels que le sang contaminé ou les essais nucléaires dans le Pacifique, l’État a commis une faute qui doit être réparée. Or le code civil est clair : l’auteur d’un dommage à autrui est tenu de le réparer. Ce principe simple et républicain ne peut être plus longtemps ignoré. Aimé Césaire nous a mis en garde : « Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Aussi, faisons preuve de courage politique, de justice et d’équité en votant ce texte. La parole

problèmes de fertilité, naissances prématurées, malformations congénitales, risque accru de cancer de la prostate chez les hommes, difficultés et retards sur le développement moteur et cognitif, tels sont les effets du chlordécone sur la santé humaine.

Cette pollution a également entraîné d’importantes conséquences économiques dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation d’abord, avec la contamination de plusieurs milliers d’hectares de terres, notamment dans la région Sud Basse Terre, en Guadeloupe, dans le secteur de la pêche, grandement impacté par la réduction de ses zones d’activité ou par les arrêtés d’interdiction visant à lutter contre l’apport de poisson contaminé. Ce scandale sanitaire, environnemental, économique et politique, avec les lenteurs, dérogations et hésitations des pouvoirs publics vis à vis de la toxicité avérée de la chlordécone, a évidemment nourri une profonde défiance des populations antillaises envers l’État et l’exigence, plus que légitime, d’une reconnaissance de la responsabilité de ce dernier et de réparations pour le préjudice subi. Le 11 mars 2025, soit dix huit ans après le dépôt de la première plainte contre la pollution au chlordécone aux Antilles, la cour d’appel de Paris a reconnu la responsabilité partagée de l’État sur l’autorisation délivrée pour sa commercialisation et son épandage dans les Antilles. Il est désormais avéré que l’État a failli dans ses missions de contrôle, d’autorisation de délivrance, de vente et d’homologation du pesticide. C’est pourquoi le texte présenté aujourd’hui, qui vise à reconnaître légalement la responsabilité de l’État et la création d’un régime juridique permettant à toutes les victimes, et non plus seulement aux professionnels exposés au chlordécone, de demander une indemnisation intégrale de leur préjudice, est évidemment regardé favorablement par le Enfin, se pencher de nouveau sur le scandale du chlordécone offre l’occasion de rappeler plus largement que les produits que nous autorisons dans nos champs, dans nos pépinières, sur nos terres, mais aussi dans la construction, peuvent présenter des risques sanitaires et environnementaux lourds, dont les impacts socio économiques sont majeurs

La protection de nos filières sur chacun de nos territoires passe par la mémoire des leçons du passé. Faut il le rappeler : prudence est mère de sûreté. Notre vote doit ainsi servir à entériner la prise de conscience par les pouvoirs publics de la pollution au chlordécone et à résorber la crise de confiance entre l’État, ses services déconcentrés, les collectivités et les associations qui alimente l’exigence de réparation pour les pour les populations des Antilles. C’est pourquoi la réponse de l’État doit marcher sur deux jambes, indissociables l’une de l’autre : une exigence de vérité et de clarté vis à vis des Guadeloupéens et des Martiniquais, et une exigence d’action concrète et ambitieuse répondant au préjudice écologique, économique et sanitaire issu de cette pollution. La parole

L’emploi du chlordécone dans les Antilles entre 1972 et 1993 est un scandale sanitaire avéré, voire un scandale d’État, tant la responsabilité de ce dernier ne fait aucun doute. Notre collègue Théophile, auteur de la proposition de loi, l’a rappelé : dès le début, l’État savait, il ne pouvait ignorer. Les faits sont là, têtus et glaçants. Dès 1968, la commission interministérielle d’études sur les pesticides avait explicitement exclu l’usage du chlordécone en raison de sa grande persistance et de sa toxicité. fut pourtant autorisé par cette même commission en 1972, alors seulement pour un an et à titre dérogatoire, pour lutter contre le charançon de la banane. Nous connaissons bien le provisoire qui dure, en voici un exemple caractéristique d’année en année, l’autorisation fut reconduite, durant vingt ans, alors que, dans le même temps, les preuves scientifiques du danger que ce produit présentait pour la santé ne cessaient de s’accumuler, chaque fois plus accablantes. Comment a t on pu reconduire l’autorisation d’usage du chlordécone alors que les États Unis eux mêmes, qui ne sont pourtant pas vraiment connus pour être un parangon de vertu sanitaire, n’y avaient plus recours depuis le milieu des années 1970 ? Comment a t on pu ignorer le rapport Snegaroff de 1977 et le rapport Kermarrec de 1980 ? Ce qui a été toléré dans les bananeraies des Antilles n’aurait sans doute jamais été accepté dans les vergers d’Occitanie ou dans les vignobles de Bourgogne. C’est incompréhensible et révoltant.

agronomique (Inra) l’a d’ailleurs explicitement déclaré : tous les milieux sont contaminés, les sols comme les eaux. Je rappelle que l’on interdit la pêche trop près des côtes pour des raisons sanitaires, que les tubercules comme l’igname ou le dachine, qui constituent une part substantielle du régime alimentaire des populations antillaises, sont des racines et sont donc contaminés. Face à ce scandale, les dispositifs d’indemnisation existants sont largement insuffisants. Aujourd’hui, seuls les travailleurs de la banane ayant développé un cancer de la prostate, ou leurs enfants exposés, peuvent être indemnisés. Et encore, les conditions d’ouverture de ces droits sont restrictives pour les travailleurs, il faut avoir été exposé au moins dix ans au produit ; pour les enfants, il faut être atteint de pathologies particulièrement graves – troubles du système nerveux, leucémie, malformation congénitale. De plus, l’indemnisation est non pas intégrale, mais forfaitaire. de remédier à ces insuffisances notoires, pour ne pas dire choquantes, la proposition de loi de notre collègue Théophile pose le principe de la reconnaissance pleine et entière de la responsabilité de l’État et crée un régime général d’indemnisation. Ce n’est pas la première fois que l’État choisit de créer ce type de régime : nous l’avons fait pour les victimes de l’amiante, pour celles des essais nucléaires et pour les enfants victimes de la Dépakine. À chaque fois, l’ampleur du dommage et l’évidence de la faute l’exigeaient. Pourquoi refuserions nous cette reconnaissance aux populations antillaises ? Pourtant, ce texte a été rejeté par notre commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. Notre rapporteure Nadège Havet, dont je salue l’investissement sur ce dossier difficile et particulièrement épineux, a développé les arguments de la commission ayant conduit à ce rejet argument de principe – l’État ne serait pas seul responsable, les industriels le sont aussi – ; argument scientifique – à l’exception du cancer de la prostate, il n’existerait pas de consensus liant exposition au chlordécone et autres pathologies argument technique – comment articuler le fonds créé par le texte avec le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides ? comment sanctionner juridiquement le préjudice d’anxiété ? – ; enfin, évidemment, argument budgétaire – en l’absence d’étude d’impact, nous ne savons pas combien coûterait le régime d’indemnisation proposé.

une énième tentative infructueuse d’avancer sur ce dossier. Nous ne pouvons plus continuer à empiler les propositions de loi et les rapports d’information sur le sujet. Aussi, nous nous en remettons aujourd’hui au Gouvernement, véritable juge de paix en pareille circonstance, pour trouver une solution qui satisfasse les aspirations légitimes des populations à la reconnaissance de leur souffrance et à la réparation de leur préjudice, dans des conditions techniques, juridiques et budgétaires cadrées pour l’État. Sur la base d’un consensus qui se dégagerait des amendements gouvernementaux, le groupe Union Centriste votera cette proposition de loi. La parole est à M. Robert Wienie Xowie.

Pourtant, l’État français a maintenu l’autorisation de vente durant treize années encore, avant de la retirer en 1990 – enfin, pas vraiment, puisque la vente a perduré trois ans de plus là où le chlordécone était le plus utilisé, en Guadeloupe et en Martinique. 77 % des travailleurs agricoles de la banane ont été directement exposés au chlordécone à l’époque où ce pesticide était utilisé. Si les professionnels sont particulièrement touchés, la réalité est que 92 % des Martiniquais et 95 % des Guadeloupéens sont contaminés, d’après les chiffres de Santé publique France. L’exposition au chlordécone a des effets connus : un risque de naissance prématurée, des conséquences sur la croissance et le développement neurologique des enfants, et un risque augmenté de cancer de la prostate.

Depuis 2020, un fonds d’indemnisation existe, mais 200 dossiers seulement ont été déposés jusqu’à présent, dont 154 ont été validés, et toutes les indemnités ne sont pas encore versées. Ce fonds est donc très insuffisant.

Le rapport de la commission indique ainsi que « la création d’une autorité administrative indépendante – le Comité d’indemnisation des victimes du chlordécone – reviendrait à consacrer un exceptionnalisme concurrent du régime général d’indemnisation des victimes de pesticides ».

en Guadeloupe et en Martinique un produit dont on connaissait les conséquences sur la santé et sur l’environnement ! Cette proposition de loi doit réparer une injustice à laquelle nous ne saurions répondre par une injustice supplémentaire. Oui, nous devons reconnaître la responsabilité de l’État dans cette contamination à grande échelle et de longue durée ; oui, nous devons indemniser spécifiquement les victimes de ce scandale sanitaire. J’ajoute que nous devons apprendre des erreurs commises à cette époque

malgré la promesse du président Emmanuel Macron en 2017 de l’interdire dans les trois ans. Celui ci disait d’ailleurs au sujet du chlordécone en 2018 : « Ce fut aussi le fruit d’un aveuglement collectif. D’où il faut d’ailleurs tirer la force de se battre aujourd’hui contre des logiques analogues. » Le fonds d’indemnisation des victimes des pesticides a d’ailleurs reconnu en 2022 le lien entre le glyphosate et les malformations. Combien de personnes faudra t il encore indemniser pour en arrêter la vente ? La santé et l’environnement doivent être une priorité ; la justice aussi. C’est pourquoi l’ensemble de notre groupe

carences et négligences fautives, action tardive, manquement au devoir d’information des citoyens, insuffisante vigilance, faillite dans ses missions de contrôle, grave impéritie administrative

Aussi est il indispensable d’inscrire dans la loi les premiers mots de l’alinéa 1 de l’article 1 de la proposition de loi de notre collègue Dominique Théophile. Reconnaître la responsabilité fautive de l’État

La version initiale de cette proposition de loi pose les bases ambitieuses d’un dispositif d’indemnisation à la hauteur des dommages ; elle résulte du constat de l’insuffisance du premier geste fait en 2020 avec l’indemnisation des victimes de pesticides, fruit de la mission de contrôle menée huit ans plus tôt par notre collègue Nicole Bonnefoy.

ont autorisé la vente d’un produit dont la dangerosité avait été scientifiquement établie bien avant son utilisation massive en Guadeloupe et en Martinique entre 1972 et 1993. Dès 1968 au moins, le caractère toxique et persistant du chlordécone était établi. On connaît, hélas ! cette tragique logique selon laquelle des intérêts économiques priment les droits humains et environnementaux, de l’amiante aux néonicotinoïdes, du flufénacet aux polyfluoroalkylées (PFAS). Quand tirerons nous vraiment les leçons de ces désastres ? Après le rejet global de ce texte en commission la semaine dernière, nous avions, hélas ! compris que son ambition serait rabotée par les amendements de la rapporteure et du Gouvernement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je remercie notre collègue Dominique Théophile d’avoir mis en débat ce texte important et attendu. Le chlordécone fait partie des pesticides organiques de synthèse à base de chlore,

Le chlordécone a fait l’objet de nombreuses études scientifiques démontrant sa toxicité neurologique et reproductive chez l’homme et chez l’animal. Ces propriétés en font un perturbateur endocrinien, notamment pour les femmes. Dans mon rapport sur les pesticides en 2012, j’indiquais que l’étude Karuprostate montrait très clairement que l’exposition au chlordécone multipliait par 1,8 le risque de développer un cancer de la prostate chez les hommes ayant une concentration en chlordécone dans le sang supérieure à un gramme par litre. Le pire dans cette substance est sa longévité. Le chlordécone n’est malheureusement pas digéré par la nature. Sa structure moléculaire se dégrade en métabolites qui n’atteignent leur demi vie qu’au bout de 46 ans et ne disparaissent totalement qu’après plusieurs centaines d’années. Le dernier rapport de l’Opecst, en mars 2023, rend compte de la première étude Kannari, conduite en 2013 et 2014, qui démontre que le chlordécone était détecté chez plus de 90 % des adultes antillais. Sur la base de ces prélèvements, il a été estimé que 14 % des adultes guadeloupéens et 25 % des adultes martiniquais dépassaient la valeur toxicologique de référence interne définie par l’Anses. Si nous voulions bien entendre ces faits, documentés dans des rapports parlementaires, nous pourrions peut être réexaminer

Le drame du chlordécone vient nous rappeler qu’en voulant être sourds aux alertes de nos agences sanitaires et scientifiques, nous prenons des risques inconsidérés pour l’environnement et la santé humaine.

un pas en avant, deux pas en arrière ! J’ai du mal à comprendre la logique. Les sols ont une meilleure mémoire que les hommes. On récolte ce que l’on sème ce vieil adage paysan est plus vrai que jamais, y compris en matière de produits phytosanitaires. En témoigne la persistance du chlordécone, dont on retrouve des traces dans les produits alimentaires locaux patates douces, ignames, mais aussi crustacés et poissons, alors même qu’ils n’ont pas même été traités par ce produit. Face à la rémanence de cette substance, le présent texte vise à reconnaître la responsabilité de l’État dans l’autorisation et l’usage du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique

par la volonté du Gouvernement d’en réduire la portée, puisque seules les maladies professionnelles sont éligibles à cette indemnisation et que cette dernière est forfaitaire et non intégrale.

compte tenu du scandale sanitaire et environnemental que représente le chlordécone, nous soutiendrons l’article 1 de ce texte, qui crée un régime spécifique d’indemnisation des victimes. Cette mesure est de nature à répondre à une situation vécue comme un scandale en Guadeloupe et en Martinique, une situation qui génère un sentiment de défiance à l’égard de l’État et de ses institutions. Ce texte permettrait de reconstruire cette confiance perdue et résoudrait les difficultés d’adhésion aux dispositifs et aux recommandations émises par les services de l’État. Cette proposition de loi vient donc donner corps à un engagement présidentiel non tenu. Elle est, par ailleurs, conforme à un récent arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Celle ci reconnaît les fautes commises par l’État, qui a autorisé la vente de ce pesticide, et demande la réparation du préjudice moral d’anxiété des personnes durablement exposées à cette pollution. Mais c’était sans compter des amendements de dernière minute, déposés par la rapporteure et le Gouvernement, visant notamment à retirer du texte la reconnaissance

Cela me rappelle fortement les débats que nous avons eus lors de la création du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides dont j’ai pris l’initiative en 2018. Si ces amendements étaient adoptés au cours de cette séance, nous aboutirions à une version moins disante

De 1972 à 1993, le chlordécone, insecticide efficace contre les parasites nuisibles aux cultures dans les bananeraies, a été largement utilisé dans les plantations de la Guadeloupe et de la Martinique. Cette molécule, largement diffusée après l’ouragan David de 1979, qui avait ravagé les plantations, plantations, s’est instillée dans les cours d’eau et les terres de ces îles, mais surtout dans le corps de nos compatriotes des Antilles. On estime que près de 90 % de la population de ces territoires est contaminée par le chlordécone, perturbateur endocrinien violent qui cause de nombreux cancers, des malformations et des difficultés reproductives. Malgré une connaissance précoce de sa dangerosité, le chlordécone n’a été interdit qu’en 1993 ; en attendant, il aura, pour des décennies, si ce n’est des siècles, pollué les terres et les eaux et détruit de nombreuses vies.

forte consommatrice de produits phytosanitaires, colonne vertébrale de l’économie de ces îles. Le chlordécone et ses effets sont un scandale. Comme dans de nombreux territoires, dont le mien, les pollutions héritées d’activités agricoles ou industrielles passées ou présentes représentent des drames économiques, sanitaires et sociaux trop grands. Du bassin minier du Pas de Calais aux bananeraies de Basse Terre, l’État doit prendre sa responsabilité dans l’indemnisation des collectivités et, surtout, des personnes touchées par les effets de ces substances. La tragédie du chlordécone illustre aussi, s’il le fallait encore, l’abandon structurel des territoires ultramarins. L’absence de toute politique réelle d’autonomie et de souveraineté, le faible développement de circuits économiques et productifs sains, voilà les phénomènes indirects et cachés qui entourent le scandale du chlordécone. Quelle économie de la mer, quelle autonomie alimentaire, quelle production antillaise propre peuvent répondre aux besoins de la population ? Tout cela, l’État n’y a jamais pourvu ; il a plutôt laissé perdurer sans contrôle, avec l’aide des forces économiques qui lui sont liées, une culture de la banane assise sur la diffusion d’un poison. Ce texte va selon nous dans le bon sens, mais nous regrettons les trop nombreux amendements dévoilés Il appartient en effet à l’État de réparer, dans les limites déjà raisonnables posées dans le texte initial, les dommages subis par les populations du fait de la diffusion massive du chlordécone. Pour autant, nous soutiendrons ce texte. La parole

Ce qu’il s’est passé aux Antilles apparaît aujourd’hui comme totalement inacceptable. Personne ne peut affirmer le contraire : utiliser pendant vingt ans un produit dont plusieurs rapports attestaient, dès l’origine, la dangerosité pour la santé humaine et l’environnement n’est pas excusable. Aucun Guadeloupéen, aucun Martiniquais n’ignore ce qu’est le scandale du chlordécone, mais, pour nos autres compatriotes, de quoi parle t on exactement ? Le chlordécone est un pesticide qui a été utilisé dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe entre 1972 et 1993. Il permettait de lutter contre le charançon du bananier, qui sévissait alors dans les plantations.

dans les bananeraies, ont été directement en contact avec le produit. Non, on parle de la quasi intégralité des habitants : 92 % des Martiniquais et 95 % des Guadeloupéens, évidemment à des niveaux de contamination différents.

y est plus de deux fois supérieur à celui que connaît l’Hexagone. Les enfants exposés au chlordécone sont exposés à des risques de pathologies du système nerveux, de leucémies et de malformations congénitales. On parle donc bien de conséquences dramatiques pour des milliers de personnes, sur plusieurs générations. On ne peut pas se dédouaner d’un phénomène qui relève non pas d’une catastrophe naturelle, mais bien d’une décision administrative, ou plutôt d’une succession de telles décisions. En effet, lorsqu’il a été autorisé pour la première fois en France en 1972, le chlordécone ne l’a été qu’à titre temporaire, pour une seule année. Cette autorisation a ensuite été renouvelée tous les ans. Même lorsque le produit a finalement été interdit en France, en 1990, une dérogation a encore été accordée pour les Antilles jusqu’en 1993 Même les États Unis avaient interdit l’utilisation et la production du chlordécone dès 1976, précisément à cause de sa toxicité. En France, sa « grande persistance » et sa « toxicité » avaient été reconnues dès 1968,

ce n’est certainement pas uniquement à l’État qu’a bénéficié l’usage du chlordécone aux Antilles pendant vingt ans. La responsabilité est évidemment partagée entre une multitude d’acteurs, y compris locaux. C’est l’équilibre complexe auquel nous sommes régulièrement soumis dans le cadre de nos débats : la nécessité de préserver une économie, derrière laquelle se trouvent des emplois et des familles, l’avancée des connaissances scientifiques, et les éventuelles conséquences sur la santé et l’environnement. La production de la banane aux Antilles est précaire. À l’instar de beaucoup de cultures hexagonales, elle est confrontée aux difficultés liées au climat, aux parasites, au non renouvellement des générations d’exploitants et à la concurrence de producteurs étrangers qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes.

Pour les victimes, qui sont des milliers de personnes, les préjudices sont évidemment réels ; quand le lien de causalité avec le chlordécone est établi, elles méritent réparation.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite d’abord saluer l’initiative de mon collègue Dominique Théophile. En déposant cette proposition de loi, il a porté haut la voix de celles et ceux que l’on n’a pas voulu entendre pendant trop longtemps. C’est un acte politique fort, un acte de justice, un acte d’espoir ! Je prends la parole aujourd’hui avec une émotion particulière, car le drame du chlordécone n’est pas un fait divers local c’est un désastre sanitaire, écologique et humain qui a durablement marqué la Guadeloupe, la Martinique et, plus largement, la Caraïbe. Le chlordécone, ce n’est pas une erreur : c’est un poison dont la toxicité était connue. Pourtant, son usage a été autorisé, prolongé, toléré. Ce n’est donc pas seulement une imprudence : c’est une faute Aujourd’hui encore, les terres sont polluées pour des siècles. L’eau, les aliments, les corps portent la trace d’une contamination invisible, mais omniprésente. Les enfants naissent avec l’angoisse héritée de leurs parents. Et, dans cette angoisse, il y a aussi le sentiment d’avoir été abandonné. Face à cela, la reconnaissance de la responsabilité de l’État est essentielle, non pas pour raviver les blessures, mais à l’inverse pour commencer, enfin, à les panser. Elle est la condition de toute réparation, de toute réconciliation. Je veux ici exprimer ma solidarité caribéenne. Même si Saint Martin n’a pas connu l’usage du chlordécone, je me tiens aux côtés de nos frères et sœurs guadeloupéens et martiniquais. L’histoire de la Caraïbe est une histoire de combats communs et, dans ce combat là, nous devons faire front ensemble. Cette proposition de loi pose des bases nécessaires : reconnaissance, indemnisation, information, prévention. Elle ne réglera pas tout. Mais elle dit à ceux qui souffrent : la République vous voit, la République vous croit, la République vous doit ! Enfin, il nous reviendra de transformer ces paroles en actes : pour réparer, dans la mesure du possible, pour garantir que cela ne se reproduira plus et pour rendre enfin justice aux victimes de ce scandale environnemental et sanitaire. Pour toutes ces raisons, je voterai sans réserve cette proposition de loi. Bravo ! La parole Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me permets d’intervenir dans cette discussion générale en tant que président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et

rapport étudiait en détail les caractéristiques particulières de cette molécule, sa grande stabilité et ses faibles possibilités de dégradation, allant jusqu’à la qualifier d’« alien chimique

la contamination des sols, des eaux fluviales, des nappes phréatiques et des milieux marins était une réalité persistante, nécessitant, d’une part, qu’une cartographie complète et détaillée de la pollution soit établie et, d’autre part, que des recherches soient activement menées sur les méthodes de dépollution. Parallèlement, des études épidémiologiques commençaient seulement à se mettre en place pour suivre la santé des populations les plus exposées et évaluer, par exemple, la possibilité d’une plus forte prévalence du cancer de la prostate, ou de problèmes neurologiques chez les nouveau nés.

À l’Opecst, nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ces recommandations aurait eu une vraie portée pour les populations de Guadeloupe et de Martinique. C’est pourquoi, monsieur le ministre, je souhaiterais que vous nous indiquiez si, au cours des dernières années, certaines de ces préconisations ont pu être mises en œuvre. J’ai déposé plusieurs amendements sur cette proposition de loi. Deux d’entre eux, malheureusement, ont été déclarés irrecevables. Je voudrais les évoquer brièvement, car, certes, les populations de Guadeloupe et de Martinique sont les premières exposées à cette pollution, mais d’autres personnes qui ont séjourné pendant plusieurs années sont également susceptibles de souffrir d’une maladie liée à l’exposition au chlordécone. Il me semblait cohérent de le mentionner. À l’inverse, la demande de réparation pour les ayants droit me semble aller trop loin. Je voudrais vraiment assurer tous mes collègues de Guadeloupe et de Martinique, ainsi que nos concitoyens antillais, du soutien réel et complet que les membres de l’Opecst apportent à leur combat pour faire mieux prendre en compte les conséquences de la pollution au chlordécone. La parole

Ce sujet constitue un véritable traumatisme collectif local, qui se double d’une incompréhension de la population face aux tergiversations politiques, s’agissant tant de la reconnaissance de la responsabilité de l’État que de la prise en charge des victimes potentielles. Ma conviction est qu’il y a des sujets qui ne doivent pas

en Guadeloupe et en Martinique, de ce qui était interdit ailleurs. Je comprends toutefois que Mme le rapporteur ait voulu laisser la porte ouverte à une voie judiciaire d’indemnisation, qui permettra d’explorer toutes les dimensions de ce sujet, en réponse à ce qui reste un besoin au sein de la population traumatisée. Comment comprendre, en outre, que l’on puisse s’interroger sur la responsabilité de l’État alors que, par ailleurs, l’hypersécurité sanitaire et la culture française de la surtransposition des normes étouffent nos agriculteurs, qui demandent de desserrer l’étau normatif ? ? Enfin, comment comprendre que, alors que l’on connaissait l’interdiction américaine du chlordécone, celui ci ait été autorisé outre mer ? Le texte qui nous est présenté pose le principe de la reconnaissance de la responsabilité de l’État et ouvre la voie à une indemnisation des victimes. Je ne peux qu’adhérer à ces deux grands principes ; je considère que le texte initial a ouvert des pistes et suscité un débat très large. Les travaux préparatoires de l’examen en séance ont cependant permis une exploration de l’ensemble de ces pistes, qui nous permettra d’aboutir à un texte équilibré rendant effective la mise en œuvre des dispositions envisagées. de ce travail de recentrage et de concrétisation, que nous devons aux populations. Il est indéniable que la conscience de la contamination a été une source d’appréhension et d’anxiété pour certains publics. Pour autant, l’ériger en préjudice aboutirait à une procédure novatrice complexe, qui susciterait probablement, elle aussi, une forme de méfiance à l’égard des critères d’évaluation du caractère légitime ou non de l’anxiété de la population. La connaissance scientifique et la recherche disposent encore de marges de progression certaines. Le rapport remis en 2023 par notre ancienne collègue Catherine Procaccia sur l’impact de l’utilisation du chlordécone aux Antilles souligne bien la nécessité à la fois de poursuivre les travaux et de rétablir la confiance de la population.

sur les Antilles. La discussion générale est close. La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi.

par le juge administratif comme par le juge judiciaire, la pollution par le chlordécone est le fruit d’un aveuglement collectif qui a conduit à accepter cette situation, parce que l’État, les élus locaux et les acteurs économiques considéraient qu’arrêter le chlordécone, c’était menacer une partie des exploitations en Martinique Je suis donc favorable à cet amendement. Nous ne pourrons pas revenir en arrière, la priorité est d’aller de l’avant pour sortir du risque lié au chlordécone. Des solutions existent, cela prendra du temps, mais nous avons besoin de tout le monde. La parole

» : j’y vois un crime, un scandale d’État. Les responsabilités sont clairement établies. Je vous demande donc, monsieur le ministre, d’arrêter de parler d’aveuglement collectif quand il s’agit de responsabilités prises en toute connaissance de cause, au mépris de la santé des Antillaises et des Antillais.

L’État reconnaît sa responsabilité dans les dommages sanitaires subis par les populations de Guadeloupe et de Martinique du fait des autorisations provisoires de vente, des homologations et des autorisations d’utilisation à titre dérogatoire accordées à des produits phytopharmaceutiques à base de chlordécone et de leur usage prolongé comme insecticide agricole. » Monsieur

La séance est reprise.

Personne ne demande plus à voter ?… Le scrutin est clos.

qu’une candidature pour siéger au sein des commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic et de la proposition de loi organique fixant le statut du procureur de la République national anti criminalité organisée a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. Mes chers collègues,

l’Agence est clair : « Le recours à des drones de pulvérisation est envisagé comme une alternative pouvant présenter de multiples avantages. » Ceux ci sont de trois ordres. D’abord, les drones permettent une amélioration des conditions de travail.

qui luttent contre la cercosporiose noire. Ces derniers sont contraints à une pulvérisation depuis le sol vers le sommet des bananiers, laquelle les expose à des retombées de produits fongicides. Je ne parle même pas de la fatigue, de la chaleur et de l’épuisement physique liés à leur travail. Pour eux, l’usage de drones répond concrètement à une réalité professionnelle très difficile. Enfin, l’usage de drones permet des gains

présentant un risque faible pour la santé humaine, aux produits de biocontrôle ainsi qu’à ceux qui sont utilisés en agriculture biologique. Cette limitation est de nature à rassurer nos concitoyens et donc à favoriser une utilisation plus large de cette technologie. En troisième lieu, des mesures de gestion des risques et des conditions d’utilisation notamment l’établissement de distances de sécurité dans les zones sensibles, garantiront la santé des personnes et la préservation de l’environnement. Grâce à ces différents garde fous, ce texte est équilibré.

définit une méthode robuste, fondée sur l’évaluation scientifique des avantages manifestes du drone pour la santé et l’environnement. Elle permettra d’étendre par voie réglementaire le dispositif aujourd’hui envisagé à de nouveaux types de parcelles ou de cultures.

la pleine maîtrise des progrès scientifiques et techniques, au bénéfice de notre production comme de la santé humaine et de la protection de l’environnement. La parole est à M. le rapporteur.

phytopharmaceutiques, l’usage de drones. J’ai conscience que la transition entre l’examen du précédent texte – le sujet était particulièrement lourd pour nos compatriotes guadeloupéens et martiniquais – et celui ci n’est pas forcément des plus simples. Soyons clairs : si, dans un cas, il s’agissait de reconnaître la responsabilité de l’État et d’indemniser les victimes du chlordécone, il est à présent question d’améliorer la protection des applicateurs de produits phytopharmaceutiques et même de réduire, à terme,

de moderniser le cadre législatif applicable à l’usage de drones pour la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques. En cela, nous continuons notre action de « désurtransposition » de notre droit national, comme d’autres pays l’ont fait avant. pays l’ont fait avant. Ce sujet est loin de nous être inconnu : nous nous sommes d’ores et déjà prononcés par deux fois dans cet hémicycle sur la question des drones en agriculture. Par deux fois, le Sénat a soutenu, dans le respect du cadre européen, une évolution de notre droit en la matière. En premier lieu, nous l’avons fait à l’occasion du vote, en mai 2023, de la proposition de loi pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, portée par nos collègues Laurent Duplomb, Pierre Louault et Serge Mérillou. fait tout récemment à l’occasion du vote, en janvier dernier, de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, déposée par nos collègues Laurent Duplomb et Franck Menonville.

Du reste, tel est le souhait de l’essentiel des acteurs agricoles que j’ai entendus dans le cadre de mes auditions. Que contient précisément cet article unique que je vous invite à adopter sans modification ?

Bien entendu, cet usage est encadré et limité. Nous ne parlons pas d’utiliser des hélicoptères pour arroser sans discrimination toute une zone avec des produits classés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

Il permettra naturellement à davantage d’agriculteurs de bénéficier s’ils le souhaitent de cette technique et donc de sécuriser l’intervention des applicateurs.

Rappelons que, en 2023 encore, la viticulture détenait le triste record d’accidents du travail graves non mortels ainsi que d’accidents du travail mortels. Si le drone est loin d’être l’alpha et l’oméga de la sécurité au travail, travail, il aide à réduire à la fois l’exposition aux produits phytopharmaceutiques et les risques d’accident liés à l’utilisation de machines agricoles dans des conditions difficiles. Nous pouvons tous nous accorder à dire que c’est un progrès. En matière d’exposition des applicateurs, je ne peux pas ne pas dire un mot de la filière de la banane. Je sais que l’usage de produits phytopharmaceutiques dans les bananeraies est une question sensible, pour des raisons dont nous venons de débattre dans le cadre du précédent texte

pour atteindre les feuilles de la cime de l’arbre et ainsi lutter contre la cercosporiose noire. Je sais que certains d’entre vous auraient souhaité adopter des dispositions spécifiques. Pour cette raison, je considère ce texte comme un point de départ : il n’épuise pas le sujet de la réduction de l’exposition des applicateurs.

Ce mécanisme permet de faire évoluer les règles de façon plus agile que si nous devions repasser par le Parlement, filière par filière, ce qui n’aurait naturellement aucun sens.

notre vote de la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. La principale différence entre le texte qui nous est soumis le dispositif précédemment adopté réside dans le pourcentage minimal de pente nécessaire à l’autorisation de l’épandage par drone : alors qu’il était de 30 %, il est désormais établi à 20 %. Ce chiffre semble tout à fait pertinent, comme l’indiquait M. le rapporteur Cabanel. Il permettra à davantage d’agriculteurs de bénéficier de cette innovation. Ce débat permet surtout de rappeler à quel point cette proposition de loi semble vertueuse pour l’évolution de notre agriculture et de notre sécurité alimentaire. Il est nécessaire de revenir sur la surtransposition au fondement de ce texte en permettant, comme les autres pays européens, d’utiliser l’innovation qu’incarnent les drones lorsqu’elle présente des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications terrestres. Cette technologie n’en est qu’à ses prémices, mais ce texte enverra un signal fort à la recherche et à l’innovation. D’abord, l’innovation est ainsi mise au service de la réduction non seulement de l’exposition des opérateurs, mais aussi de la quantité globale de produits phytopharmaceutiques et d’eau utilisés. elle est mise au service de l’attractivité du métier d’agriculteur par la réduction des contraintes et de la pénibilité, alors que se profile le mur du renouvellement des générations. Enfin,

rédaction proposée est un compromis, équilibré et proportionné : la protection tant de l’individu que de notre environnement est prise en compte. Les dispositions de ce texte permettent d’améliorer les conditions de travail sans porter atteinte à nos acquis en matière en matière environnementale puisque son champ est circonscrit à l’épandage de produits à faible risque ou autorisés en agriculture biologique. L’Anses conservera la responsabilité d’évaluer les avantages et les risques de cette méthode. En effet, cette levée de l’interdiction de principe ne suffit pas à autoriser les pulvérisations de produits phytopharmaceutiques par drone : il restera nécessaire d’étendre à un usage aérien les autorisations de mise sur le marché des produits concernés.

ces essais « doivent être considérés avec précaution compte tenu du jeu de données très restreint ». Aussi, « l’analyse des données ne permet pas, à ce stade, de dégager des conclusions générales robustes compte tenu des incertitudes observées

envoyons un signal positif à la recherche et à l’innovation tout en accompagnant nos agriculteurs, dans l’attente d’une technologie qui permettra l’identification des maladies sur pied, afin de les traiter dès la première infection.

Ce postulat relève de l’évidence pour bon nombre d’entre nous dans cet hémicycle. Pourtant, je sais que les débats seront une nouvelle fois nourris ce soir. Sans revenir en détail sur l’histoire de ce texte,

À l’issue de cette expérimentation, l’Anses a rendu un rapport d’évaluation et conclu que le recours à des drones de pulvérisation représente une « alternative pouvant présenter de multiples avantages et l’environnement (Inrae) a également conclu à une plus grande efficacité de cette technique. Toutefois, l’expérimentation étant arrivée à son terme, il n’est plus autorisé de réaliser des pulvérisations par drone en France, là où le droit européen offre des marges de manœuvre. Nous nous retrouvons donc – encore ! – en situation de surtransposition, cette fois ci involontaire : les drones ne faisaient pas partie du débat lorsque nous avons établi cette interdiction stricte en transposant la directive SUD () en droit interne. Néanmoins,

Alors, pourquoi tant d’engouement pour ces engins volants ? Eh bien, imaginez : un drone pèse moins qu’un pulvérisateur dorsal de quarante kilogrammes, ne se renverse pas sur une pente raide et, surtout, n’expose pas de la même manière les travailleurs aux produits pulvérisés. Je reprends les mots de l’Anses : « Les résultats indiquent que l’exposition de l’opérateur utilisant un drone est environ 200 fois plus faible que pour un opérateur utilisant un chenillard. C’est donc une bénédiction pour les agriculteurs, qui gagnent en confort, en sécurité et probablement en espérance de vie. Ces drones sont aussi écolos ils réduisent les phénomènes de dérive, car la pulvérisation se fait beaucoup plus proche du sol. Leur précision permet de mieux cibler les traitements et de moins utiliser de produits.

Rappelons également que la légalisation de l’utilisation de ces nouvelles technologies est un enjeu de souveraineté alimentaire puisque notre capacité à produire Les acteurs des différentes filières sont demandeurs : à nous de leur offrir une solution pérenne et équilibrée ! Nos voisins l’ont d’ailleurs bien compris puisque l’Allemagne, l’Autriche ou encore la Belgique se sont saisies des dérogations offertes par l’Union européenne pour autoriser ces pratiques. posons – c’est normal ! – un cadre strict. Le texte ne concerne que trois catégories de produits : produits de biocontrôle, produits autorisés en agriculture biologique et produits à faible risque. Nous levons l’interdiction de principe seulement dans trois cas lorsque la pente est supérieure ou égale à 20 %, pour les bananeraies et pour les vignes mères de porte greffes, rares, mais essentielles au renouvellement Cela étant, si l’expérimentation permise par ce texte, qui étend les programmes de pulvérisation par drone des mêmes produits à d’autres types de parcelles et de cultures, est évaluée favorablement par l’Anses, il sera nécessaire d’étendre en conséquence le régime d’autorisation.

mes chers collègues, pour assurer le développement durable de notre agriculture, nous avons besoin de promouvoir toutes les modernisations, donc de soutenir toutes les recherches tendant à l’optimisation des outils et des process de production, surtout quand il s’agit de limiter la consommation de produits phytosanitaires, d’économiser l’eau et de réduire au maximum les gaspillages ! C’est la raison pour laquelle nous soutenons les missions de recherche de l’Inrae, prenons en compte les expertises produites par l’Anses et soutenons les politiques publiques dont l’objectif est de pérenniser les spécificités de notre agriculture familiale en ne laissant aucune ferme sur le bord de la route. Nous choisissons cette option, car nous savons qu’il n’y a pas de ruralité vivante sans agriculteurs ! Monsieur le rapporteur, je tiens à saluer l’excellence de votre approche. En votre qualité de professionnel de la viticulture ayant choisi la conversion au bio, vous vous montrez extrêmement sensible à la qualité des produits agricoles et à la protection de la santé des agriculteurs,

qui vous revendiquez pleinement comme héritier des philosophes des Lumières ! Merci de nous avoir rappelé combien le progrès des sciences et des techniques peut améliorer les conditions de production,

liminaire – que la mécanisation motorisée de l’agriculture est encore minoritaire à l’échelle mondiale. La traction animale reste très présente et la traction humaine, principalement assurée par des femmes, demeure utilisée dans quelques contrées du monde. lors, quand l’occasion se présente de déployer des technologies nouvelles pour servir la cause du mieux être de l’humanité, il ne faut pas s’en priver ! Et, avec vous, j’ai envie de dire à mon tour : « Vive le progrès ! Mais le progrès ne vaut que par les usages qu’il procure. Et on sait bien qu’il y a un abîme entre le silex et l’énergie cosmique. Piloter l’étincelle du silex pouvait être à la portée de chacun. Piloter l’énergie cosmique implique d’autres règles, quelques connaissances – pardonnez moi – et quelques précautions ! Tel est aussi le cas du pilotage des drones et de leur utilisation pour épandre des produits phytopharmaceutiques. La culture viticole étant faiblement développée en Bretagne, je me garderai bien de tout commentaire sur les avantages attendus du développement de cette pratique. Très sensible aux désastres produits par l’épandage du chlordécone – nous en avons parlé tout à l’heure –, je me garderai bien aussi de critiquer les avantages légitimes attendus de cette technique.

difficiles à conjuguer et à coordonner ! Plus la loi s’oblige à entrer dans le détail et la précision, plus elle devient précaire et contestable.

de loi s’inscrit dans le prolongement de la loi Égalim de 2018, qui avait remis en cause le principe de l’interdiction absolue de l’épandage aérien de pesticides. Alors que le monde agricole traverse une crise sans précédent, faute de politiques publiques garantissant des prix rémunérateurs pour nos paysans, alors que le système de l’agrochimie altère tous les pans de notre biodiversité, il nous paraît clair, à nous, écologistes, que pérenniser l’utilisation de drones pour la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques n’était pas une priorité – c’est peu de le dire

permettent d’améliorer les conditions de travail des agriculteurs, dans le respect de la santé humaine et environnementale. Mais il paraît assez évident qu’en l’espèce de telles conditions ne sont pas réunies. collègues, vous vous limitez à autoriser les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle et les produits autorisés en agriculture biologique, et ce sur quelques types de parcelles seulement, mais nous craignons qu’il ne s’agisse là que d’un cheval de Troie, destiné à enterrer, à terme, le principe de l’interdiction des pulvérisations aériennes

quand il faudrait procéder à une évaluation objective de l’ensemble des incidences au lieu de produire des données partielles et orientées. Au travers de cette proposition de loi se pose également la question de notre modèle agricole. Ah ! Ce texte ouvre la voie à la généralisation de l’usage des drones, il alimente l’endettement et un système productiviste à bout de souffle… Oh là là ! … et il lève peu à peu les obstacles à des usages renouvelés des pesticides, alors que les efforts devraient porter sur la recherche et le déploiement de solutions alternatives, pour engager enfin une véritable transition agroécologique. L’usage de technologies importées crée d’ailleurs une réelle dépendance et obère notre souveraineté.

Au passage, je suis surpris – c’est un faible mot – de la juxtaposition dans cette niche de deux textes pour le moins contradictoires. D’une part, il est question – ou plutôt il était question – de reconnaître la responsabilité de l’État dans l’utilisation du chlordécone en Guadeloupe et en Martinique. Je prends acte, au demeurant, que la majorité sénatoriale ne nous a pas permis de le faire. C’est ça, oui… Je vous remercie de valider mes propos, ma chère collègue ! D’autre part, et c’est pour le moins surprenant, il est question de réautoriser l’épandage comme si la réalité des scandales sanitaires du passé n’avait aucun effet sur la façon dont nous légiférons aujourd’hui. Ce principe général d’interdiction de la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques, on le doit à une directive européenne d’octobre 2009, adaptée en droit français la loi du 12 juillet 2010

Surtout, et c’est bien là le plus important, l’Anses ne donne aucun avis tranché et préconise plutôt de poursuivre les expérimentations avant d’envisager une quelconque généralisation, « dans la mesure où les études montrent des résultats pouvant présenter une forte variabilité ».

On en revient inévitablement, comme toujours, à la logique productiviste, commerciale et compétitive. Nous sommes conscients qu’il existe une véritable problématique liée à la spécificité de certains territoires, et particulièrement des territoires ultramarins. Aussi ce sujet mériterait il que soit ouverte une réflexion spécifique pour que des aménagements puissent être trouvés, dès lors que toutes les garanties de sécurité pour l’homme et pour l’environnement seraient réunies. Pour être tout à fait clair quant à notre position, il convient de dissocier la technique visée, d’une part, et les produits utilisés, d’autre part. Jamais les socialistes ne refuseront le progrès, et surtout pas quand celui ci vise à améliorer les conditions de travail. L’usage d’un drone en tant que tel ne nous pose donc pas de problème En revanche, jamais nous ne défendrons l’usage des pesticides. Jamais nous ne dirons aux paysans : « Utilisez des pesticides ; les rendements de cette année seront meilleurs, mais dans trente ans votre santé en pâtira. L’enjeu n’est donc pas celui de la technologie : il y va bien de la santé des paysans, des consommateurs, des riverains, des sols, de la faune, de la flore, des milieux aquatiques. Notre position n’a jamais changé : nous avons toujours été hostiles à l’épandage aérien de pesticides.

épandus des espaces situés à proximité de la zone d’épandage. La dérive lors des épandages aériens est d’autant plus importante que le vent est fort. » Ce rapport, qui fut adopté à l’unanimité, prônait l’application stricte du principe de précaution, ce dont la proposition de loi que nous examinons

Il est certain que l’avenir est à l’emploi d’automates de toutes sortes, et les drones font clairement partie du tableau. Soyons clairs ! L’objectif n’est surtout pas le retour aux épandages à l’ancienne, par hélicoptère ou par ULM, avec toute leur imprécision. Mais ce texte ne vise pas non plus

Le principe général reste donc l’interdiction du traitement par aéronef. Ainsi ce texte prévoit il trois dérogations extrêmement encadrées, pour une ouverture que certains jugeront responsable et mesurée, quand je la trouve, personnellement, minimale et sans ambition.

nous allons continuer d’avancer vers une agriculture plus vertueuse, moins dangereuse pour l’applicateur – c’est très important – et toujours plus respectueuse de l’environnement : une agriculture attractive

je me réjouis que nous examinions, pour la troisième fois depuis 2023, un texte relatif à l’usage des drones dans l’agriculture. Comme le rapporteur l’a très justement indiqué, nous nous sommes déjà prononcés à deux reprises sur ce sujet

visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, adoptée par le Sénat il y a moins de trois mois. J’ai eu le plaisir d’être le rapporteur de ce dernier texte ; la disposition relative aux drones ne m’est donc pas tout à fait étrangère,

avec Mme la ministre, que je remercie une fois encore de son action résolue en la matière. Il est donc logique pour nous de soutenir le présent texte, qui prévoit la possibilité de déroger à l’interdiction générale de la pulvérisation aérienne, pour un usage par drone faisant l’objet d’un strict encadrement. En effet, les produits autorisés dans le dispositif proposé sont les produits homologués les moins dangereux, et les usages concernés se limitent à trois situations, à savoir les parcelles en pente, les vignes mères porte greffes et les bananeraies. L’ensemble est encadré par des dispositions réglementaires dont la charge de l’édiction reviendra notamment au ministre chargé de l’agriculture, après avis de l’Anses. Autant dire que nous sommes loin d’une ouverture incontrôlée des vannes ! Il s’agit plutôt de tirer parti des possibilités offertes par le droit européen pour permettre à notre agriculture de faire ce qu’elle a toujours fait : s’adapter et se moderniser. Cette modernisation se ferait d’ailleurs au bénéfice des applicateurs de produits phytopharmaceutiques, dont il est prouvé que l’exposition s’en trouverait significativement réduite – les conclusions de l’Anses en la matière sont parfaitement claires. Elle se ferait aussi au bénéfice de l’environnement et de la réduction de l’usage des intrants. En effet, si nous pouvons d’ores et déjà localiser par drone le développement d’adventices au sein d’une parcelle, nous pourrons demain,

La semaine dernière, à l’invitation du président du groupe d’études Agriculture, élevage et alimentation, Laurent Duplomb, nous sommes allés dans l’Oise assister à une démonstration de pulvérisation par drone d’eau sur un verger.

une fois de plus sa volonté de répondre aux attentes des professions agricoles, qui souhaitent l’adoption de ce texte. Après une expérimentation menée entre 2019 et 2022 de la loi Égalim 1, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a constaté, au gré de ses travaux, les bienfaits de l’épandage par drone.

Par ailleurs, l’épandage par drone s’avère particulièrement utile à certains types d’environnements. Je pense notamment aux zones dont les sols sont instables, comme les rizières, aux cultures dont les plantes sont ouvertes vers l’extérieur,

Je n’oublie pas non plus les vignes mères porte greffes, qui sont quasi enterrées dans le sol. L’Anses relève en outre dans sa note que « plusieurs essais d’efficacité conduits en Suisse ont […] montré que des traitements par drone pouvaient fournir une protection similaire à des traitements au sol […] en cas de faible pression en maladies sur vigne De surcroît, les drones sont légers, rapides, manœuvrables et précis. Autrement dit, dans certaines conditions biologiques, végétatives, climatiques et topographiques, l’épandage par drone est une solution intéressante, dont les avantages pour traiter plus efficacement les maladies affectant les cultures végétales et préserver la santé humaine, celle, en l’espèce, des agriculteurs. Je rappelle également que l’autorisation d’épandage, qui s’appliquera uniquement aux environnements spécifiques précédemment cités, sera strictement encadrée et limitée aux produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique et aux produits associés de biocontrôle. telles opérations devront faire l’objet, de nouveau, d’une évaluation favorable de l’Anses. Mes chers collègues, nous avons l’occasion de voter conforme un texte attendu par les professions agricoles,

pour un choc de compétitivité en faveur de la ferme France, et en janvier 2025, dans la proposition de loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. Par conséquent, notre groupe votera dans sa grande majorité pour ce texte. La parole

l’agriculture française est un pilier de notre économie et de notre patrimoine. Nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos producteurs font face à des défis croissants, comme le changement climatique, la pression économique et des exigences environnementales toujours plus strictes. Dans ce contexte, nous avons la responsabilité d’accompagner ces hommes et ces femmes qui nous nourrissent, en leur donnant accès aux outils les plus innovants. C’est précisément l’objet de cette proposition de loi, qui vise à autoriser, sous conditions strictes, l’usage des drones pour le traitement des maladies affectant les cultures végétales. Depuis 2011, la France interdit la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques, décision motivée par la nécessité de préserver la santé publique et l’environnement. Toutefois, cette interdiction généralisée a aussi ses limites. Certaines parcelles agricoles, notamment en zones pentues ou difficiles d’accès, ne peuvent pas être traitées efficacement par des moyens terrestres, mettant en péril les récoltes et la viabilité des exploitations. La présente proposition de loi ne revient pas sur l’interdiction de principe. Elle vise simplement à l’adapter aux réalités du terrain, en autorisant, dans des conditions strictement encadrées, l’utilisation d’aéronefs télépilotés pour l’épandage de produits de biocontrôle et à faible impact environnemental. Il ne s’agit donc ni d’un retour en arrière ni d’une concession aux pratiques du passé : c’est bien une avancée pragmatique, raisonnée et responsable. L’adoption de ce texte offrira plusieurs avantages majeurs à notre agriculture. Tout d’abord, elle permettra une application plus ciblée et plus précise des traitements, réduisant ainsi l’usage global de produits phytosanitaires et limitant la dérive des substances dans l’environnement. Ensuite, elle répondra à une demande forte des agriculteurs confrontés à des conditions topographiques complexes, notamment en zones montagneuses ou sur des cultures spécifiques, comme la banane et les vignes mères porte greffes. Enfin, et surtout, elle protégera leur santé. Les expérimentations récentes menées en Alsace et en Ardèche viennent renforcer cette conviction. Les résultats sont sans appel : les drones permettent une réduction significative de l’exposition des opérateurs aux bouillies de traitement, ainsi qu’une baisse des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Parmi les secteurs qui bénéficieront directement de cette évolution, la viticulture occupe une place centrale. Nos vignobles, souvent situés sur des terrains escarpés et difficiles d’accès, sont particulièrement exposés aux maladies telles que le mildiou ou l’oïdium. Aujourd’hui, les viticulteurs doivent mobiliser des moyens lourds, coûteux et parfois dangereux pour traiter leurs vignes. Les drones offrent une alternative plus sûre, plus efficace et plus respectueuse de l’environnement. Ils préservent la santé des travailleurs agricoles en réduisant leur exposition directe aux produits, limitent les risques de maladies professionnelles et d’accidents, tout en assurant une grande précision dans les traitements. Depuis 2015, en Alsace, des acteurs engagés, tels que les Domaines Schlumberger, la CFTC AGRI et la Caisse d’assurance accidents agricoles du Haut Rhin, ont démontré, par leur travail de terrain et leurs démarches auprès des autorités, que la technologie drone pouvait être mise au service de la sécurité des personnes. Il est aussi essentiel de rappeler que la directive européenne de 2009 interdisant la pulvérisation aérienne visait spécifiquement les hélicoptères et les avions. C’est par surtransposition nationale que les drones ont été inclus dans cette interdiction. Une telle interprétation n’est pas suivie par d’autres pays européens, comme l’Allemagne et l’Autriche. La Suisse, quant à elle, assimile la pulvérisation par drone à une pulvérisation au sol ; c’est vers cette définition qu’il faudrait tendre. de loi constitue non pas une autorisation généralisée, mais une adaptation nécessaire, encadrée et limitée à des situations spécifiques. En la votant, nous faisons le choix du progrès raisonné, du soutien à notre agriculture et de l’innovation au service du développement durable.

celle d’un chenillard, plusieurs études montrent, en revanche, que les dépôts sur les cultures présentent une variabilité supérieure après l’utilisation de drones qu’avec des matériels d’application classiques.

a pour vocation, demain, à généraliser l’épandage de toutes sortes de pesticides sur toutes sortes de cultures. C’est bien cela qui est en filigrane et qui adviendra dans quelques années si nous votons cet article 1. Quel est

entre, d’un côté, l’ouverture, dans certains contextes, de l’usage des drones en agriculture et, de l’autre, de vraies assurances que l’on ne peut pulvériser n’importe quoi à n’importe quel moment.

en lien avec un système de monoculture intensive qui apporte tout un lot de maladies. Et bien entendu, la réponse est alors le traitement et le surtraitement.

Cette expérimentation est justement très cadrée : elle est menée sur les bananeraies et sur des surfaces agricoles plantées en vigne et présentant une pente supérieure ou égale à 30 %, afin d’obtenir des

Nous proposons donc que l’Anses dresse un nouveau bilan d’ici à deux ans. Cette durée nous paraît suffisante pour permettre la tenue d’études complémentaires. Quel

Sept ans et une évaluation de l’Anses plus tard, je pense que nous devons aller de l’avant. Et, si je suis profondément

la pulvérisation par les drones se fait par le dessus – cela coule un peu de source ! Elle se fait sur certaines cultures lorsque le développement foliaire n’est pas important. Mais, pour certaines maladies,

L’interdiction de tout épandage aérien – par drone ou autre – pour les bananes a conduit à demander aux opérateurs de traiter par le dessous, alors que la maladie commence par le dessus.

pour traiter la cercosporiose des bananes, nous diminuerions encore l’utilisation des produits phyto à six passages. Il faudrait ne pas se poser la question de l’utilisation du drone

Cet amendement revêt pour nous une importance majeure. Il s’agit de supprimer le droit à l’essai prévu par le I de l’article 1, qui illustre concrètement les risques de dérive que nous dénonçons si la présente proposition de loi venait à être adoptée en l’état. ce droit à l’essai reviendrait, concrètement, à réautoriser l’épandage aérien de pesticides en France sur tout le territoire, et ce sans jamais avoir à revenir devant le Parlement pour en débattre. concerne toutes les cultures et toutes les parcelles, indépendamment de la présence d’un risque majeur avéré ou de topologie particulière justifiant un tel recours. Si le texte tente d’apporter certaines garanties en termes d’encadrement, nous savons très bien qu’il reviendra surtout

nous voyons bien que l’objectif est progressivement de supprimer toutes les réglementations, de réautoriser des pesticides interdits, de diminuer le pouvoir des opérateurs de l’État, comme l’Anses ou l’Office français de la biodiversité, et de procéder à un énorme retour en arrière sur le plan environnemental. Certains nous répondront que seuls certains produits sont, à ce stade, concernés par cette dérogation, ou que ce droit à l’essai ne pourra être pérennisé qu’à l’issue d’une évaluation de l’Anses, ce qui est bien le minimum. Cependant, nous considérons que le contexte politique actuel de défiance majeure à l’égard du monde scientifique et des agences fera peser bien trop de pression sur l’Anses, qui est déjà largement attaquée

par cette dérogation, certains tenteront, demain, d’en élargir la liste dès que l’occasion se présentera. Pour nous, ces alinéas illustrent parfaitement le risque de fuite en avant que susciterait l’adoption de la présente proposition de loi en l’état. Nous réaffirmons donc, par cet amendement, que le principe de précaution doit primer avant tout et que l’exception ne doit pas devenir la règle. ne doit pas devenir la règle.

Je répète, en effet, que l’expérimentation est une bonne méthode, encore plus lorsqu’elle est encadrée et contrôlée, comme dans le cas présent. Je rappelle que les expérimentations pourront effectivement être menées, mais que, si les évaluations menées par l’Anses ne sont pas concluantes, elles ne seront pas

pose un cadre, c’est au pouvoir réglementaire de s’assurer de l’application de ce cadre ! C’est exactement ce que fait ce texte : il pose un cadre et définit les règles.

en effet, la rédaction de l’alinéa que votre amendement vise reprend quasiment mot pour mot la condition essentielle à l’usage des drones figurant à l’article 9 de la directive européenne de 2009 sur les produits phytopharmaceutiques. Il n’est donc pas nécessaire de la modifier. Avis défavorable. Quel est

dérogatoire au principe général d’interdiction de la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques. Pour les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, la rédaction retenue dans le cadre de cette proposition de loi pourrait laisser planer une ambiguïté qui semble peu opportune au vu des inquiétudes que suscite par ailleurs la philosophie d’ensemble du texte. En effet, le code rural prévoit actuellement que le principe de la dérogation à l’interdiction générale d’épandage aérien, d’une part, ne peut se déclencher qu’en cas de danger sanitaire grave et, d’autre part, concerne la pulvérisation de produits destinés à lutter contre ce danger. Or la rédaction de la proposition de loi n’apporte pas cette dernière précision. Dans l’absolu, elle pourrait donc ouvrir la possibilité de recourir à l’épandage aérien en cas de danger sanitaire grave, même si les produits épandus n’ont pas vocation à spécifiquement à spécifiquement lutter contre le danger identifié. À ce titre, il semble préférable d’en rester à la rédaction actuelle de l’article L. 253 8, en vigueur depuis 2016.

Cet amendement de repli vise à bien préciser que la dérogation au principe général d’interdiction en cas de danger sanitaire grave ne peut porter que sur la pulvérisation de produits visant à lutter contre ce danger identifié.

modification de pure forme. La nouvelle formulation qui est proposée à l’alinéa 3 ne diffère que très légèrement de l’actuelle et ne change absolument rien au fond.

la rédaction de l’alinéa 4 concernant la prise en compte de la pente pouvant donner lieu à des dérogations. La rédaction actuelle prévoit que cette autorisation pourrait être donnée, à titre dérogatoire, sur des parcelles agricoles comportant une pente supérieure à 20 %. Or il est apparu que cette rédaction était sujette à interprétation, comme cela a été d’ailleurs le cas au moment des débats à l’Assemblée nationale, sans qu’une réponse très claire soit apportée en retour. En effet, le terme « comporter » pourrait laisser penser qu’une parcelle inclinée à un pourcentage inférieur à 20 %, mais comportant seulement une zone supérieure à 20 %, pourrait en bénéficier. Nous estimons bien évidemment que ce n’est pas l’esprit de la loi et qu’il s’agit bien de viser les parcelles dont les pentes sont supérieures à un pourcentage donné, qu’il soit, d’ailleurs, de 20 % ou de 30 %. Nous proposons donc d’en rester au terme utilisé actuellement dans la législation, à savoir

d’interdiction de pulvérisation aérienne de pesticides est autorisée. L’expérimentation issue de la loi Égalim 1 portait sur une pente supérieure ou égale à 30 %.

que pourrait induire cette proposition de loi si elle était adoptée en l’état. L’abaissement de ce pourcentage sans aucune étude d’impact l’illustre parfaitement. Les défenseurs de la suppression pure et simple de l’interdiction de l’épandage aérien se saisiront dès qu’ils le pourront d’un nouveau texte pour pour abaisser encore ce seuil ou pour prévoir d’autres régimes dérogatoires. Dans ces conditions, il convient d’en rester au régime d’exception.

Dans son évaluation de 2022, l’Anses indique ainsi, concernant les drones : « Les conditions d’utilisation ont un impact très important sur le niveau de la dérive. En effet, le vent, le type de buse, la vitesse d’avancement du drone et la hauteur de pulvérisation sont des facteurs ayant un impact important sur la dérive. » À ce titre, il paraît donc nécessaire de prévoir, comme c’est déjà le cas dans la réglementation en